La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 20 février 2020 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. chers collègues, j'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Michel Charasse, qui fut sénateur du Puy-de-Dôme de 1981 à 1988 et de 1992 à 2010. Un hommage lui sera rendu dans l'hémicycle par le président du Sénat la semaine prochaine.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi simplement d'un mot de dire à quel point le décès de Michel Charasse, qui fut votre collègue, mais qui fut aussi le mien au Conseil constitutionnel, m'a bouleversée. C'était un très grand républicain et, en plus, un ami très proche et très cher. Monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, cher Philippe Bonnecarrère, mesdames, messieurs les sénateurs, nous examinons donc aujourd'hui le projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée. Certains contentieux pénaux présentent, en raison de leur nature ou de leur gravité, une spécificité particulière qui justifie qu'ils fassent l'objet de règles de procédure adaptées faisant intervenir des magistrats spécialisés. C'est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour lesquelles il a paru nécessaire à plusieurs États membres de l'Union d'instituer une coopération renforcée se traduisant par la création d'un tout nouvel organe judiciaire : le Parquet européen. C'est également le cas, au niveau national, des infractions relevant de la criminalité organisée, de la grande délinquance financière, du terrorisme ou des atteintes à l'environnement, pour lesquelles existent d'ores et déjà des juridictions spécialisées, qu'il s'agisse des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS), du parquet national financier (PNF), des pôles spécialisés en matière de santé publique et d'environnement, ou encore du parquet national antiterroriste Le présent projet de loi a pour objectifs principaux d'adapter notre législation à la création du Parquet européen et d'améliorer les dispositifs actuels concernant la justice pénale spécialisée nationale. Le titre I de ce projet de loi adapte notre législation au règlement du Conseil européen du 12 octobre 2017, qui a prévu la création du Parquet européen. La création de ce nouvel organe judiciaire européen constitue une étape supplémentaire dans le développement de l'espace judiciaire européen. Du traité de Maastricht au traité d'Amsterdam, notre pays a toujours accompagné une vision engagée et volontaire de la construction de l'Union européenne et de cette Europe judiciaire. Le Sénat lui-même a été présent à chaque étape de cette longue construction. Je souhaite donc ici rendre un hommage particulier au rôle que le Sénat a joué en ce domaine. Il faut en effet rappeler que votre assemblée a historiquement soutenu le principe même de la création de ce Parquet européen, alors même que celui-ci ne paraissait être encore qu'une chimère. Plusieurs résolutions du Sénat ont ainsi appelé à la création de cet organe judiciaire, dont l'une dès 2002, avec le soutien actif de Robert Badinter, apôtre inlassable de la construction européenne. Sur ce sujet, le Sénat ne s'est pas contenté de pétitions de principe. Ainsi, lorsque la Commission européenne a déposé son projet de règlement portant création du Parquet européen, le Sénat n'a pas hésité à réaffirmer son soutien de principe, tout en portant des exigences précises sur ses modalités de mise en oeuvre. La Chambre haute a en effet adopté à l'époque une résolution portant sur le respect du principe de subsidiarité. Jointe aux résolutions de même nature émanant d'autres parlements nationaux, elle a conduit pour la première fois, dans le contexte de l'espace de liberté, de justice et de sécurité, à la procédure dite du « carton jaune ». Ce faisant, cette procédure a contraint la Commission à une réponse motivée aux griefs qui lui étaient faits de ne pas se conformer au principe de subsidiarité. Certes, à l'issue de cette procédure, la Commission a maintenu son projet initial, mais, lors du conseil Justice et affaires intérieures de juin 2014, c'est une orientation générale en faveur d'un Parquet européen collégial, disposant d'une compétence concurrente à celle des autorités nationales, qui a été dégagée. Le « carton jaune » n'y a pas été totalement étranger. Le règlement du 12 octobre 2017 doit donc beaucoup au Sénat, et je me réjouis de vous présenter aujourd'hui le projet de loi qui assure la compatibilité entre notre droit interne et les équilibres issus du texte de l'Union. Le Parquet européen s'inscrit dans le cadre d'une coopération renforcée, qui réunit à ce jour 22 États membres sur les 27 de l'Union. Si l'on excepte l'Irlande et le Danemark, qui bénéficient de régimes dérogatoires en matière de coopération judiciaire et policière, ce projet réunit donc en réalité 22 États sur 25. Seules manquent à l'appel la Suède, la Pologne et la Hongrie. La Suède a déjà annoncé son intention de rejoindre le projet ; concernant la Pologne et à la Hongrie, je suis certaine qu'à long terme ils y viendront ... Permettez-moi de dire maintenant quelques mots du Parquet européen. Celui-ci sera compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des fraudes qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union, à savoir les escroqueries à la TVA, les faits de corruption, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance, de blanchiment d'argent, ainsi que certains délits douaniers. Le schéma retenu permet d'assurer un juste équilibre entre, d'une part, part, l'efficacité de la répression contre une délinquance astucieuse qui est largement internationale et dont les profits se chiffrent parfois en millions d'euros, et, d'autre part, la préservation de l'autonomie et de la souveraineté de notre ordre judiciaire, puisque les juges du tribunal judiciaire de Paris demeureront compétents pour juger ces infractions et, le cas échéant, condamner leurs auteurs aux peines prévues par le code pénal français. Le Parquet européen siégera à Luxembourg, capitale judiciaire de l'Union. Il sera dirigé par un procureur européen, en la personne de Laura Kövesi, qui sera assistée de 22 procureurs nationaux- un par État membre participant. Le Parquet européen comportera aux échelons nationaux des procureurs européens délégués chargés, dans chaque État, du suivi des enquêtes et des poursuites. Ils seront au minimum deux par État. Pour ce qui concerne la France, ils seront à Paris. Afin de permettre à ces procureurs européens délégués français d'exercer leur mission, le projet de loi- c'est évidemment cela qui est important -modifie le code de procédure pénale, le code de l'organisation judiciaire et le code des douanes. Ces modifications ont pour objet premier de leur garantir une totale indépendance. Ils ne pourront recevoir d'instructions que du Parquet européen ils ne pourront donc pas recevoir d'instructions générales du ministre de la justice ni même d'instructions générales ou particulières du procureur général de Paris. Les modifications proposées procèdent par ailleurs aux adaptations procédurales nécessaires pour permettre à ces procureurs européens délégués français de conduire leurs investigations et d'exercer des poursuites devant les juridictions françaises. Il est ainsi prévu que ces procureurs européens délégués disposent des mêmes prérogatives que le procureur de la République, ainsi, et c'est beaucoup plus novateur, que certaines prérogatives relevant de la compétence du juge d'instruction. Ils pourront ainsi placer un individu sous contrôle judiciaire ; ils pourront, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention (JLD), placer des suspects sous écoutes téléphoniques ; ils pourront également solliciter l'autorisation du JLD pour placer un suspect en détention provisoire. Ce dispositif est donc très novateur dans notre procédure pénale puisqu'il confie au procureur délégué européen des pouvoirs aujourd'hui exercés par des juges d'instruction. Mais c'est le règlement du Parquet européen qui le prévoit et ce dispositif n'a pas vocation à être perçu comme une première étape d'évolution de notre droit interne vers la suppression du juge d'instruction. Ces dispositions, qui devraient entrer en application avant la fin de l'année 2020, permettront d'améliorer de manière significative la lutte contre les fraudes aux intérêts de l'Union. Je me réjouis que votre rapporteur et votre commission des lois, dont je veux ici souligner la qualité du travail, aient accepté ces dispositions en les améliorant sur certains points techniques. Le titre II du projet de loi est relatif à la justice pénale spécialisée. Il consolide l'efficacité et la cohérence des dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la délinquance organisées, la délinquance économique et financière. loi tend également à assurer un traitement contentieux plus efficace des atteintes à l'environnement. Concernant les juridictions spécialisées, en premier lieu, le texte prévoit de faciliter l'exercice des compétences des parquets spécialisés afin de mieux prendre en considération leur expertise et les objectifs qui avaient présidé à leur création. Il est ainsi prévu que les parquets spécialisés pourront, en cas de compétences concurrentes avec d'autres parquets, exercer leurs compétences prioritairement par rapport aux parquets non spécialisés. Ce dispositif permettra aussi de résoudre les conflits de compétences de manière efficace. En deuxième lieu, le titre II procède à une extension des compétences du parquet national antiterroriste, qui pourra notamment représenter le ministère public aux audiences d'assises de première instance en matière de crimes contre l'humanité, de crimes de tortures et de disparitions forcées, de crimes et délits de guerre. Il reconnaît par ailleurs une compétence concurrente à ce même parquet national antiterroriste pour certains crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation. En troisième lieu, ce même titre II renforce les compétences du parquet national financier afin d'assurer la meilleure efficacité possible en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, en lui conférant, en la matière, une compétence nationale concurrente. Sur le point spécifique de la lutte contre les atteintes à l'environnement, le projet de loi hisse notre organisation judiciaire à la hauteur de notre ambition politique et des attentes de nos concitoyens en matière de contentieux environnemental. La justice tient un rôle incontournable de régulation en prévenant, en sanctionnant et en réparant les atteintes écologiques. Pourtant, aujourd'hui, le contentieux environnemental représente seulement 1 % des condamnations pénales et 0,5 % des condamnations civiles. Ces chiffres ne reflètent pas pour autant la réalité des atteintes qui sont portées quotidiennement à l'environnement et à la biodiversité. Ils ne rendent pas davantage compte de l'activité des services de l'État chargés du respect de la réglementation applicable. L'action quotidienne des inspecteurs de l'environnement permet, par la mise en oeuvre des mesures de police administrative, de prévenir, de sanctionner, voire de réparer les infractions les plus courantes à l'égard de l'environnement. Mais certaines atteintes exigent une réponse judiciaire effective et plus rapide, car ces actes constituent des dommages graves et irréversibles à l'environnement pour lesquels une réponse administrative ne peut suffire pour faire cesser les manquements. Aussi, lorsque la justice est saisie, elle doit être efficace. Cela passe par une organisation et des réponses judiciaires rénovées. Nous créons donc dans ce texte une justice pour l'environnement construite en première instance sur trois niveaux. Pour la préservation du cadre de vie de nos concitoyens, nous confortons une justice de proximité. Je pense aussi aux affaires qui concernent la vie quotidienne des Français et des élus locaux : par exemple, les décharges sauvages, les permis de construire illégaux, les infractions à la réglementation sur la pêche ou la chasse, la pollution visuelle et sonore. et sonore. Ces affaires seront jugées par les tribunaux judiciaires dans chaque département. Quand plusieurs tribunaux judiciaires existent dans un même département,

Pour la protection contre les atteintes graves ou la mise en péril de l'environnement, nous créons une juridiction spécialisée de première instance par ressort de cour d'appel. Ces juridictions pour l'environnement auront vocation à traiter, par exemple, les pollutions d'effluents ou des sols par des activités industrielles, les infractions au régime des installations classées qui dégradent l'environnement, les atteintes aux espèces ou aux espaces protégés, les infractions à la réglementation sur les déchets industriels, etc. Nous spécialisons dans ce cas-là à la fois les magistrats qui dirigent ces enquêtes et ceux qui jugeront les affaires. Cela permettra de raccourcir le délai de traitement des procédures, qui, actuellement, n'est pas satisfaisant. Cela permettra aussi de mieux maîtriser la technicité du droit applicable. Enfin, dernier étage, pour les accidents industriels causant des victimes multiples ou pour les risques technologiques majeurs- je pense ici aux activités nucléaires nous maintenons les pôles nationaux environnement et santé publique qui existent aujourd'hui et qui sont basés à Paris et à Marseille. Ils sont compétents à eux deux sur l'ensemble du territoire national. Typiquement, une affaire comme celle de Lubrizol restera de la compétence de l'un de ces pôles. Quelle que soit la juridiction de première instance saisie, les affaires seront évidemment jugées en appel par la cour d'appel territorialement compétente. Nous apportons également avec ce texte des réponses judiciaires rénovées. au-delà de cette nouvelle organisation judiciaire que je viens de vous présenter, il est indispensable, me semble-t-il, de relever le niveau des réponses judiciaires. Si vous l'acceptez, nous allons donc créer une nouvelle réponse judiciaire plus rapide, ciblant la réparation du préjudice occasionné et responsabilisant les entreprises : il s'agit de la convention judiciaire écologique. Il n'est plus acceptable qu'il soit économiquement rentable pour une entreprise de causer un préjudice écologique ou de s'affranchir des règles qui permettent de préserver notre santé et notre cadre de vie. Le dispositif de la convention judiciaire écologique est inspiré de la convention judiciaire d'intérêt public, qui est déjà utilisée dans la lutte contre la corruption et la fraude. Face aux risques encourus par l'entreprise d'une procédure judiciaire longue entraînant la mise en cause des dirigeants et une grave détérioration de son image, la démarche consiste à instaurer une procédure coopérative efficace entre la personne morale et l'autorité judiciaire. Elle permettra, sous le contrôle du juge, la réparation du préjudice en complément du versement d'une amende. Cette réponse est particulièrement adaptée aux atteintes portées à l'environnement, car elle permet de mettre rapidement en place des mesures de réparation environnementale ou/et un programme de mise en conformité. Elle est également intéressante en ce qu'il s'agit de responsabiliser les entreprises et de les mobiliser sur l'importance des enjeux écologiques, et non de rechercher seulement la responsabilité pénale des dirigeants.

en matière d'environnement et de développement durable pour les particuliers qui commettent des petites infractions portant atteinte à l'environnement. C'est ce que nous appelons les « TIG verts ». J'ai demandé au directeur de l'Agence du travail d'intérêt général d'en faire l'un de ses axes de développement, en liaison avec les associations, les collectivités locales et les départements. Ces dispositions découlent de la loi de réforme pour la justice. Je souhaitais les évoquer, car elles permettent de dresser un panorama complet de la réponse pénale qui peut être apportée aux délits environnementaux.

Le titre III du projet de loi comporte plusieurs dispositions diverses, essentiellement en matière pénale. Celles-ci ont notamment pour objet de compléter certaines dispositions de simplification de la procédure pénale, qui résultaient de la loi du 23 mars 2019. À la suite

peuvent, en vertu d'une autorisation générale du parquet, faire procéder à des examens médicaux et psychologiques. Il permet aux OPJ de faire procéder, sans autorisation du parquet, à des comparaisons d'empreintes ou de traces génétiques ou digitales. Les modifications proposées tirent également les conséquences de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) récentes du Conseil constitutionnel. Le code de procédure pénale est tout d'abord modifié pour permettre aux jurés d'assises d'être pleinement éclairés sur l'existence et le fonctionnement de la période de sûreté, dans le cas où ce dispositif serait attaché de plein droit à la peine prononcée par la cour. Ce même code est ensuite modifié pour permettre aux prévenus placés en détention provisoire en matière criminelle depuis plus de six mois de s'opposer à ce que les audiences devant la chambre de l'instruction se tiennent par visioconférence, de sorte qu'ils puissent, le cas échéant, comparaître physiquement. ensuite à instituer, au sein du code des transports, une nouvelle peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les réseaux de transports publics. Elle pourra être prononcée contre les contre les personnes ayant commis des infractions graves ou répétées dans les transports en commun. Il s'agit de la reprise d'une disposition censurée par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier dans la loi d'orientation des mobilités.

Enfin, le projet de loi comportait une habilitation à mettre en place, par ordonnance, un dispositif de péréquation et d'aide à l'installation sur l'ensemble du territoire pour les professions de notaire, d'une part, d'huissier de justice d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, d'autre part. Il s'agissait de pérenniser et de généraliser les dispositifs de péréquation déjà mis en place par ces deux professions,

de substituer à cette habilitation un mécanisme qui conforte les dispositifs existants au sein de chacune de ces deux professions, tout en assurant un droit de regard des pouvoirs publics sur ceux-ci. L'amendement adopté vise ainsi expressément à attribuer au Conseil supérieur du notariat et à la Chambre nationale des commissaires de justice la faculté de percevoir des contributions volontaires obligatoires pour financer les aides à l'installation ou au maintien des professionnels. L'objectif initial du recentrage du dispositif de péréquation et d'aide à l'installation sur ces professions est ainsi préservé, et l'objectif de la loi de 2015, respecté. Les conséquences sur le périmètre du fonds interprofessionnel d'accès au droit et à la justice pourront être précisées dans le cadre de de la navette parlementaire, en concertation avec les professionnels concernés. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, en dépit de son apparence technique, ce projet de loi présente une importance politique particulièrement significative en ce qu'il permet à la France de se conformer à un engagement européen qu'elle a porté avec force et conviction ces dernières années, à savoir la création du Parquet européen. Par ailleurs, ce texte permettra d'améliorer singulièrement le fonctionnement de notre justice pénale pour le traitement des contentieux spécialisés les plus complexes, que j'ai évoqués devant vous, particulièrement en matière d'atteintes à l'environnement, ce qui constitue un point extrêmement important. Je vous demande ainsi de bien vouloir adopter ce texte, en étant persuadée qu'il recueillera auprès de vous une très large adhésion. La parole

22 pays - ce sujet a été traité dans le cadre d'une coopération renforcée -désignera un représentant ; la collégialité fixera les règles du jeu.

et de la détention français qui examinera les choses, avec l'exercice d'une voie de recours devant la chambre d'instruction de Paris. Enfin, la juridiction française, ou plus exactement parisienne, traitera les dossiers,

en tant que procureur et le poursuivra, si des actes techniques plus précis sont nécessaires, en qualité de juge d'instruction, d'où le statut hybride, évoqué par Mme la garde des sceaux,

priorité à la juridiction spécialisée sur celle de droit commun et à la juridiction de niveau national sur celle qui exerce à l'échelon territorial. Cette position n'a fait l'objet d'aucune difficulté, qu'il s'agisse des syndicats de magistrats ou des avocats.

Merci

Entre le détournement de fonds européens, la fraude à la TVA, la corruption ou encore le blanchiment d'argent, ce sont, chaque année, plusieurs dizaines de milliards d'euros qui échappent au budget de l'Union européenne et de ses États membres. Cela a notamment pour conséquence de mettre en péril leur capacité à lever de l'argent et à mettre en oeuvre leurs politiques économiques et sociales, ainsi que la confiance des entreprises et des citoyens européens dans leurs institutions. À titre d'exemple, selon une étude publiée en septembre 2019, la Commission européenne estime à 137 milliards d'euros les pertes de recettes de TVA en 2017. La fraude en serait la principale explication. Quant à la fraude aux fonds européens, le rapport de notre collègue Patrice Joly, rendu en juillet dernier, faisait état d'un manque à gagner de plus de 390 millions d'euros pour l'Union européenne. Il faut rappeler que ces statistiques sont à nuancer. Tout d'abord, ces opérations sont par nature difficiles à évaluer ; ensuite, parce que fondées sur les signalements effectués par les États membres, sont bien souvent le reflet de leur volonté ou de leur capacité à détecter la fraude. En raison du préjudice évident pour l'Union européenne, il était indispensable de mettre en place un effort de répression concerté et conjoint, afin de garantir une protection effective de ses intérêts financiers. C'est la raison pour laquelle, sur le fondement de l'article 86 du traité de Lisbonne et sous l'impulsion de notre pays et de l'Allemagne, 22 pays de l'Union européenne ont signé, le 12 octobre 2017, le règlement mettant en oeuvre une coopération renforcée et instituant un Parquet européen. Cette nouvelle autorité judiciaire viendra compléter l'arsenal constitué de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), d'Eurojust, d'Europol et des parquets nationaux. L'ordonnance relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal constituait une première étape vers ce renforcement de la lutte contre la fraude au niveau européen. Ce mouvement est aujourd'hui poursuivi par la mise en place du futur Parquet européen, qui siégera à Luxembourg fin 2020 et sera compétent pour enquêter sur et poursuivre les infractions pénales portant atteinte au budget de l'Union européenne. Le présent texte prévoit d'adapter les procédures et l'organisation judiciaires à la création de cette nouvelle autorité judicaire, afin d'éviter les problèmes de concurrence de compétences avec d'autres juridictions nationales spécialisées, notamment le parquet national financier. Il dote les deux procureurs européens délégués, agissant au niveau déconcentré, de pouvoirs importants. L'intégralité des prérogatives des magistrats du parquet leur sont confiées, leur indépendance

Par ailleurs, le procureur européen délégué pourra ordonner des placements sous contrôle judiciaire, soumis au recours du JLD, puis, le cas échéant, à celui de la chambre de l'instruction. de faire face aux nouveaux types de délits, le projet de loi comporte également des dispositions traitant de la justice pénale spécialisée, qui tantôt renforcent les compétences de ces juridictions- c'est le cas pour celles qui sont spécialisées dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la délinquance organisées, la délinquance économique et financière -, tantôt créent de nouvelles juridictions spécialisées au sein de chaque cour d'appel- ainsi des nouveaux pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes graves à l'environnement. Le projet de loi prévoit, pour ce dernier contentieux, une réponse pénale adaptée, en permettant au procureur de la République de conclure, sur le modèle de de la transaction pénale et tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, une convention judiciaire environnementale avec une personne morale mise en cause, convention qui imposerait à cette dernière Dans tous ces domaines, en cas de concurrence de compétences et tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, la priorité sera accordée au parquet bénéficiant d'une compétence spécialisée. Le groupe La République En Marche soutient avec force les efforts déployés collectivement pour lutter avec détermination contre la fraude et la corruption au sein de l'Union européenne. Nous saluons également la volonté du Gouvernement de faire en sorte que la justice soit rendue plus rapidement, par des magistrats spécialisés, et nous félicitons de ce qu'un effort particulier ait été réalisé pour renforcer l'efficacité de la réponse pénale en matière de lutte contre les atteintes à l'environnement.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, ce projet de loi est porteur, selon nous, d'au moins deux projets de loi importants : l'un sur le Parquet européen, l'autre sur la justice environnementale. Mais ce n'est pas tout. Vous l'avez dit : d'autres sujets viennent s'agréger à ces deux volets principaux,

fait, de surcroît, à grand renfort d'ordonnances- vous savez ce que nous en pensons -et de procédure accélérée, afin de traiter en un temps record des sujets aussi techniques que disparates. J'en viens au fond du projet. Premièrement, concernant le Parquet européen, sa mise en place est l'aboutissement de longues négociations, de près de dix ans, entre l'Union et ses États membres. Le projet originel de Parquet européen « très intégré » avait fait l'objet de vives critiques, en particulier du Sénat français,

Pour notre part, nous y sommes plutôt favorables. Si le nombre d'affaires dont se saisira, ou dont sera saisi, le Parquet européen semble assez limité- les procédures concernées seront, en France,

Cependant, la création de ce parquet ne va pas sans soulever, à nos yeux, quelques questions. Qu'en est-il, d'abord, de la garantie d'indépendance promise aux parquetiers européens ? Le procureur mènera seul l'intégralité des investigations en matière d'atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, et exercera les poursuites devant le tribunal judiciaire de Paris. « Si son indépendance est reconnue par le règlement, elle risque pourtant de rester une chimère si elle n'est pas entourée de garanties », estime le Syndicat de la magistrature. Or le projet reste muet sur les conditions de cette indépendance, le Gouvernement expliquant avoir fait le choix d'une mise à disposition du magistrat français souhaitant exercer ces fonctions. Aussi la cohérence entre le statut de ce Parquet européen, en situation de détachement, et celle du parquet français actuel pose-t-elle question. La création du Parquet européen aurait pu être l'occasion d'envisager une réforme en profondeur du statut des magistrats du parquet, réforme que nous demandons depuis longtemps. À cet égard, madame la garde des sceaux, qu'en est-il du projet de réforme tant attendu sur le sujet ? Très bien ! Par ailleurs, le procureur européen délégué pourra, à son appréciation, mener l'enquête selon les règles applicables à l'enquête parquet ou selon les règles applicables à l'instruction, en se passant du juge d'instruction. Cela pose aussi question, d'autant que les compétences du parquet, pour l'instant limitées aux affaires financières, pourront ou pourraient par la suite être étendues, notamment en matière d'antiterrorisme. Nous serons vigilants sur ce point, sachant en outre que cette extension de l'arsenal judiciaire de l'Union européenne

du contrôle aux frontières et d'une fermeture aux extracommunautaires, modèle d'ailleurs largement inefficace pour enrayer la criminalité transfrontalière, qu'il s'agisse de terrorisme, de trafic de drogue ou d'immigration clandestine. J'en viens au volet environnemental du projet. Afin de remédier à la grande faiblesse du contentieux environnemental, l'article 8 institue une convention judiciaire d'intérêt public en matière environnementale, qui concernera les personnes morales. Désengorger les tribunaux par le recours à la justice « transactionnelle », d'inspiration américaine, ne nous laisse présager rien qui vaille : sans la tenue d'un procès en bonne et due forme et avec des droits de la défense inexistants, ces conventions ne permettront pas une reconnaissance explicite de la culpabilité de l'auteur du délit.

Pour notre part, nous considérons qu'il est urgent de donner davantage de crédit à la justice environnementale et, surtout, d'accorder de vrais moyens aux polices de l'environnement. Or les moyens des agences de l'État, que ce soit l'Agence française pour la biodiversité ou l'Institut

Si, en vertu de la dimension « pédagogique », soulignée en commission par M. le rapporteur, nous pouvons partager l'avis de Greenpeace, qui considère que « ces juridictions spécialisées permettraient aux magistrats d'être plus à l'aise avec les dossiers environnementaux », nous ne pouvons cependant que regretter l'insuffisance, voire l'inutilité- des juridictions spécialisées, en effet, existent déjà -, des dispositifs proposés par le Gouvernement pour répondre à cette question essentielle pour les décennies à venir. Enfin,

depuis de nombreuses années, les règles de notre procédure pénale ont été adaptées afin de mieux régler certains contentieux pénaux spécifiques dont, en raison de leur nature ou de leur gravité, le traitement justifiait des procédures particulières faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisés. Cette spécialisation fut engagée en 1986 en matière de lutte contre le terrorisme, cette lutte justifiant de donner une compétence nationale spécialisée aux aux juridictions parisiennes, puis poursuivie par la création de nombreuses autres compétences spécialisées, au niveau national ou interrégional, notamment en matière économique et financière, de délinquance et de criminalité organisées, de santé publique ou de crime contre l'humanité. Cette exigence de spécialisation a plus récemment conduit à la création du parquet national financier par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique puis du parquet national antiterroriste par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Cette exigence de spécialisation a également conduit à l'adoption du règlement européen du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, afin d'améliorer la lutte contre les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Les principaux objectifs du projet de loi que nous examinons cet après-midi sont ainsi d'adapter notre législation à la création du Parquet européen et de poursuivre l'amélioration des dispositifs actuels de notre droit national concernant la justice pénale spécialisée. Ce texte appelle plusieurs remarques. En premier lieu, la création du Parquet européen s'inscrit dans la perspective de la construction d'un espace européen de liberté, de sécurité et de justice. de respecter la souveraineté des États en matière judiciaire, son organisation est cependant décentralisée : les procureurs européens délégués, désignés dans chaque État membre, seront chargés de conduire les enquêtes et de représenter le ministère public devant les juridictions de jugement nationales. Cette organisation décentralisée n'était pas celle qui avait été envisagée par la Commission européenne lorsque celle-ci avait présenté, en 2013, sa proposition initiale de règlement portant création du Parquet européen. Ce projet de la Commission était, à l'origine, très intégré : un procureur unique aurait disposé d'une compétence exclusive pour mener des enquêtes dans toute l'Union européenne. Ce projet s'est heurté à la ferme opposition de plusieurs États membres. En effet, pour la première fois, 14 chambres parlementaires nationales, dont le Sénat français, ont mis en oeuvre la procédure dite du « carton jaune »- rien à voir avec le football -, estimant que la proposition de la Commission européenne ne respectait pas le principe de subsidiarité. Après quatre années de négociation, je me réjouis qu'un compromis ait été trouvé autour de quelques principes : compétence partagée avec les autorités nationales ; organisation collégiale ; désignation de délégués nationaux chargés de conduire les enquêtes dans chaque État membre. Ce compromis n'a toutefois pas convaincu la totalité des États membres de l'Union européenne, ce qui a justifié de recourir à la procédure dite de coopération renforcée. 22 États, à l'exclusion de l'Irlande et du Danemark, qui bénéficient d'une clause dite d'« » dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, ainsi que de la Hongrie, de la Pologne et de la Suède, qui ont refusé de s'y joindre. ce projet de loi, dans son titre II, étend les compétences des parquets nationaux spécialisés, prévoit la création d'un pôle spécialisé dans le contentieux environnemental dans le ressort de chaque cour d'appel, d'appel, et fixe des règles destinées à régler les conflits de compétences entre juridictions. Ces dispositions ne présentent aucune difficulté.

la création d'une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les réseaux de transport public et une demande d'habilitation du Gouvernement à définir par ordonnance les modalités de financement d'un fonds destiné à favoriser une présence équilibrée sur le territoire des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.

Elle a également complété les dispositions relatives à l'interdiction de paraître dans les transports publics, pour rendre cette mesure opérationnelle. Elle a en outre supprimé la demande d'habilitation que je viens d'évoquer, afin d'autoriser directement les ordres professionnels des commissaires de justice et des notaires à percevoir, auprès de leurs membres, des contributions destinées à financer des aides à l'installation ou au maintien des professionnels. À cet égard, je tiens à saluer la qualité des travaux du rapporteur, notre collègue Philippe Bonnecarrère. Madame la ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants porte un regard positif sur ce texte, d'autant que la structure du Parquet européen, dans sa conception actuelle, est une victoire du Sénat français ! Il votera donc ce projet de loi à l'unanimité.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le 17 juillet 2013, la Commission européenne a déposé une proposition de règlement afin de créer un Parquet européen, avec l'intention de « combler les lacunes du système répressif actuel, qui repose exclusivement sur les efforts nationaux, et d'assurer une plus grande cohérence et une meilleure coordination de ces efforts ». Or, en la matière, il y a bel et bien urgence à agir. Je rappelle que, entre 2010 et 2017, l'Office européen de lutte antifraude a recommandé le recouvrement de plus de 6,6 milliards d'euros pour le budget de l'Union européenne. Il a par ailleurs présenté plus de 2 300 recommandations concernant des mesures judiciaires, financières, disciplinaires et administratives que devraient prendre les autorités compétentes des États membres et de l'Union européenne. Je rappelle également que l'Office européen de lutte antifraude ne dispose d'aucun pouvoir de sanction. La Commission européenne estime quant à elle que la fraude à la TVA pourrait, à elle seule, représenter près de 50 milliards d'euros de pertes par an pour les budgets des États membres de l'Union européenne. Il n'est pas inutile de rappeler aussi que ce projet de règlement a d'abord été rejeté par de nombreux États membres, dont la France, puisqu'il s'appuyait sur l'idée de créer un Parquet européen incarné par un procureur unique et disposant d'une compétence exclusive pour enquêter sur et poursuivre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Cette première proposition s'opposait donc directement au principe de subsidiarité. À l'issue de nombreuses négociations, c'est finalement en ayant recours au mécanisme de la coopération renforcée que les ministres de la justice français et allemand de l'époque ont fait avancer le texte, l'idée d'une coopération collégiale sous la forme de procureurs délégués. Le règlement a été définitivement adopté le 12 octobre 2017, et le nouveau Parquet européen reposera sur deux organes distincts d'une part, le collège, composé d'un chef du Parquet européen et de procureurs européens ; d'autre part, des chambres permanentes, mises en place par le collège, qui superviseront et dirigeront les enquêtes en décidant notamment des classements sans suite, des procédures de poursuites simplifiées ou des renvois des affaires devant les juridictions nationales. L'un des enjeux principaux est donc de donner au procureur délégué des compétences qui relèvent en France du seul juge d'instruction. Le projet de loi donne compétence au procureur européen délégué pour recourir à des actes qui relèvent normalement du juge d'instruction. Il pourra placer la personne mise en cause sous contrôle judiciaire mais ne pourra pas prendre seul des mesures attentatoires aux libertés comme l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le placement en détention provisoire. Seul le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur européen délégué, sera compétent pour autoriser ces mesures- Enfin, l'ensemble des affaires seront jugées par les juridictions parisiennes, à savoir le tribunal judiciaire et la cour d'appel. Comme le souligne notre collègue Philippe Bonnecarrère, que je salue, dans son favorablement accueilli par notre commission des lois, ne peut que satisfaire l'ensemble de nos concitoyens. Le Parquet européen a également le mérite de rassembler l'ensemble des services de l'Union européenne, que ce soit l'Office européen de lutte antifraude ou l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs. En effet, Europol pourra être amené à fournir toute information pertinente au sujet des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, et à apporter une aide à l'analyse dans le cadre d'une enquête. enquête. Je note également que ce projet de loi permettra de mieux traiter les infractions environnementales, madame Assassi, puisque trois quarts des procédures aboutissent à des alternatives aux poursuites. D'ailleurs, la durée des procédures a un impact direct sur les sanctions prononcées, qui n'apparaissent pas toujours dissuasives et à la hauteur des enjeux environnementaux. Selon l'étude d'impact, sur 1 993 personnes sur 1 993 personnes physiques condamnées en 2018, seules 27 ont écopé de prison ferme et 954 se sont vu infliger des amendes fermes d'un montant de 1 464 euros en moyenne. Sur 139 personnes morales condamnées en 2017, il n'y a eu que 60 amendes fermes. Le Parquet européen permet donc de renforcer la construction d'une justice européenne qui permettra à l'Union de se défendre efficacement contre les atteintes à ses propres intérêts. Selon l'étude d'impact, le Parquet européen devrait récupérer entre 60 et 100 dossiers français par an. Je salue également le souhait du Gouvernement de faire figurer dans ce projet une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports publics.

Paris, le nombre de vols à la tire ait progressé de 40 % entre 2018 et 2019. Pas moins de 31 000 infractions de ce type ont été recensées dans le métro parisien. Chacun sait qu'elles sont le plus souvent commises par des multirécidivistes dont le visage est parfaitement connu des forces de l'ordre sur le terrain, ainsi que du personnel de la RATP. Celui-ci joue d'ailleurs un rôle extraordinaire de prévention, que je salue, en alertant régulièrement les passagers.

cela aurait été compréhensible. Le Sénat, comme vous l'avez souligné, a beaucoup travaillé sur le sujet. Or ce texte vise à mettre en oeuvre en France ce règlement européen, auquel nous adhérons.

la mise en oeuvre d'un système permettant de poursuivre les atteintes aux intérêts de l'Union paraît bonne. C'était une attente de la commission. Il est logique que le procureur existe pour envisager des poursuites, mais il n'y a pas d'atteinte à la souveraineté des États.

Nous avons pensé que vous pourriez, en tant que garde des sceaux, être sensible à la question de l'accès au droit et à la justice. Pour l'accès au droit et à la justice, il existe des professionnels, auxiliaires de justice, qui sont les avocats.

tant que l'État n'aura pas réglé le problème de la juste rémunération desdits avocats en matière de commission d'office et d'aide juridictionnelle ! C'est d'ailleurs ce que vous demande en partie le Conseil national des barreaux (CNB). Nous vous proposons donc, à l'occasion de ce texte, de vous exprimer en tant que garde des sceaux, garant du bon fonctionnement de la justice. Vous savez qu'à l'heure actuelle la justice ne fonctionne pas bien

de survivre ! Le précédent président du CNB nous disait que les avocats gagnent bien leur vie quand ils font du droit des affaires et du conseil. Le jour où il n'y aura plus d'avocats prêts à assurer les commissions d'office et l'aide juridictionnelle,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi dont nous discutons aujourd'hui comporte des dispositions très variées, plus ou moins attendues par nos concitoyens. L'adaptation de notre système judiciaire à l'instauration d'un Parquet européen, en particulier à l'installation de procureurs délégués dans chaque État membre, vient clore un long processus de négociations européennes. Le groupe du RDSE ne peut que saluer la mise en oeuvre d'une nouvelle coopération renforcée au sein de l'Union européenne. Cela devrait permettre d'accroître la lutte contre les fraudes portant préjudice aux intérêts financiers de l'Union, et donc des citoyens européens. Certains considèrent que cette réforme pose une nouvelle fois la question de l'avenir de la procédure pénale en France et des places respectives du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ainsi que du juge d'instruction dans cette procédure. Je laisserai aux juristes de cet hémicycle- ils sont nombreux -le soin d'expliquer pourquoi ces évolutions nécessitent de mener à bout l'indépendance du parquet. Bien qu'elles concernent la qualité de la justice rendue et l'autorité de la loi, il n'est pas certain que ces questions fassent partie des préoccupations premières de nos concitoyens. Au contraire, d'autres mesures du texte touchent plus directement à leurs préoccupations contemporaines. Je pense à la multiplication des juridictions spécialisées, souvent localisées à Paris, qui semble s'inscrire à contre-courant du grand besoin d'accessibilité aux services publics. Les quelques amendements que nous avons déposés pour délocaliser certains de ces magistrats dans des ressorts provinciaux visent à ouvrir le débat. Je pense Je pense également aux attentes en matière de protection de l'environnement, qui sont elles aussi de plus en plus partagées au sein de notre société, ne serait-ce que lorsqu'elles sont nécessaires pour préserver la santé publique. La décision du tribunal administratif de Lyon du 26 septembre 2019 ayant reconnu une faute de l'État à raison des insuffisances du plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération lyonnaise répond à la demande de réparation du préjudice d'une mère pour elle et son enfant. De fait, nos concitoyens se tournent de plus en plus vers la justice pour que leur droit à vivre dans un environnement sain soit respecté. Madame la ministre, je voudrais donc d'abord saluer l'inscription d'un titre consacré à la justice pénale environnementale dans ce texte. J'y vois une réponse à la promesse faite par votre collègue Brune Poirson dans ce même hémicycle il y a un peu moins d'un an, au moment de l'examen de la proposition de loi sur l'écocide. Je crois en effet que la voie pénale ne doit pas être écartée pour prévenir la pollution de notre écosystème. À cette fin, vous proposez l'instauration de pôles régionalisés spécialisés et le recours à la convention judiciaire d'intérêt public, mais je crains qu'il ne s'agisse d'avancées quelque peu ambivalentes et insuffisantes.

vous appelez « TIG verts », pour l'insertion sociale par des peines utiles à la société. Il y a une vingtaine d'années, lorsque j'étais maire de la commune de Saint-Nolff, c'est avec plaisir que j'ai chaque fois joué le jeu des travaux d'intérêt général.

d'amendements destinés à explorer d'autres pistes. En matière pénale comme dans les autres champs des politiques publiques, la prise de conscience écologique rebat toutes les cartes. L'éparpillement des infractions visant à sanctionner des atteintes à l'environnement

devraient être considérablement renforcés. Il comporte plusieurs pistes d'améliorations civiles et administratives qu'il aurait été utile d'intégrer, ce que l'article 45 de la Ces considérations me semblent prioritaires par rapport à la nécessité d'instaurer une nouvelle peine complémentaire d'interdiction d'utiliser les transports publics, que l'on comprend mal.

à nos amendements. En conclusion, je citerai le sociologue philosophe Bruno Latour : « Ce monde me va tout à fait, je n'en connais pas de meilleur ; d'ailleurs, je n'en ai pas d'autre.

la protection des personnes et des biens requiert que notre organisation judiciaire soit en phase avec un monde où les échanges se multiplient sans considération des frontières, y compris quand ces échanges sont le fait de réseaux criminels bien organisés. Le projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui entend, dans cet objectif, adapter la législation française à la coordination nécessaire avec le Parquet européen et à renforcer l'efficacité de la justice pénale spécialisée. C'est une joie pour moi de voir enfin arriver ce texte en séance. En effet, fin 2012, je rendais un rapport au nom de la commission des affaires européennes du Sénat, favorable à la création du Parquet européen et, le 15 janvier 2013, le Sénat votait déjà une résolution en ce sens. L'organisation du Parquet telle qu'elle est conçue par le règlement vient en grande partie de la prise de position du Sénat français. En effet, quelques mois après l'adoption de la résolution que je viens d'évoquer, notre commission recevait le projet de la Commission européenne, projet extrêmement centralisateur et directif, qui allait totalement à l'encontre de nos préconisations. Je remercie Simon Sutour, qui était alors président de la commission des affaires européennes, pour son appui et la détermination dont il a su faire preuve. La Commission européenne, faisant fi de notre souci de préserver la souveraineté et les usages des États membres, était bien décidée à imposer la création d'un parquet très intégré. Nous avons alors décidé de voter une nouvelle résolution, cette fois-ci contre ce projet, pour non-respect du principe de subsidiarité. Quatorze parlements nationaux se sont prononcés dans le même sens,

C'était une première étape. Les négociations au sein du Conseil ont finalement permis d'aboutir au règlement du 12 octobre 2017 créant le Parquet européen sous la forme d'une coopération renforcée, dans une configuration conforme aux positions françaises et aux préconisations du Sénat.

Mais la règle de l'unanimité rend cette perspective lointaine et l'excellent travail d'Eurojust réduit l'urgence. La fraude contre les intérêts financiers de l'Union européenne est aujourd'hui largement répandue, et les failles dues au manque de coordination et de coopération entre les États membres sont en grande partie responsables La Commission européenne estime que la seule fraude à la TVA représenterait 50 milliards d'euros de pertes par an pour les budgets des États membres, soit un tiers du budget de l'Union européenne. Le Parquet européen sera compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. En pratique, il pourra notamment s'agir d'escroqueries à la TVA, de faits de corruption, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance, de blanchiment d'argent et de certains délits douaniers.

Installé à Luxembourg, il comportera un bureau central composé d'un chef et de vingt-deux procureurs, soit un par État membre, et reposera sur deux organes distincts : le collège, qui assurera le suivi général des activités, la définition de la politique pénale et répondra aux questions générales soulevées par certains dossiers spécifiques ; les chambres permanentes, qui superviseront les enquêtes en décidant notamment des classements sans suite, des procédures de poursuite simplifiées ou des renvois des affaires devant les juridictions nationales. Les procureurs européens délégués (PED) représenteront, quant à eux, un échelon déconcentré au sein de chaque État et seront chargés du suivi opérationnel des enquêtes et des poursuites. Il s'agit là, à mon sens, d'une organisation respectueuse de la souveraineté des États membres, qui devrait permettre un ancrage solide dans les systèmes nationaux et être acceptée par les praticiens. Par ailleurs, ce projet de loi prévoit des dispositions relatives à la justice pénale spécialisée. Il prévoit l'exercice prioritaire de compétence en cas de ministère public spécialisé et l'extension des compétences du parquet antiterroriste, et comporte des dispositions relatives à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées, les pratiques anticoncurrentielles et les atteintes à l'environnement ; mon collègue Hervé Maurey développera ce dernier point dans quelques minutes. Ce projet de loi comporte enfin des dispositions diverses, notamment, à l'article 11, la création d'une peine complémentaire de « non-parution dans un réseau de transport public Sur ce point, monsieur le rapporteur Philippe Bonnecarrère, que je félicite pour son travail, a déposé un amendement visant à renforcer la garantie des droits de la personne condamnée. L'article 12 du projet de loi vise à tirer les conséquences des difficultés de mise en oeuvre du fonds interprofessionnel d'accès au droit et à la justice (FIADJ) institué par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui est un texte touffu. Le Parquet européen sera la première instance européenne indépendante disposant de compétences judiciaires propres. Il s'agit là d'une première étape dans la création d'un ordre public européen, nécessaire à notre unité.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, mon propos portera sur l'article 8 de ce projet de loi, la création d'un nouvel outil pour lutter contre la délinquance environnementale- la convention judiciaire d'intérêt public -et celle de pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement. madame la ministre, que cette réforme de la justice environnementale ait surgi presque inopinément, au détour d'un projet de loi technique relatif au Parquet européen, sans que les commissions parlementaires compétentes n'en aient été ne fût-ce qu'informées avant la présentation du texte en conseil des ministres, voilà moins d'un mois. On peut d'autant plus déplorer ce procédé que le Sénat a toujours été en pointe sur les questions de justice environnementale. J'évoquerai à titre d'exemple l'institution d'un régime de responsabilité du fait des atteintes à l'environnement

Sur le fond de l'article 8, l'idée de créer des juridictions spécialisées en matière d'environnement est ancienne et promue par de nombreux acteurs.

Comment espérer des résultats satisfaisants, notamment une réduction des délais, sans moyens supplémentaires ? En outre, l'essentiel du contentieux, qui touche aux sujets du « quotidien »- les décharges sauvages ou les permis de construire illégaux, par exemple -, continuera à être traité par les tribunaux judiciaires départementaux. Quant aux accidents industriels majeurs, tel celui de Lubrizol, à Rouen, ils resteront du ressort des pôles interrégionaux de Paris et de Marseille. On le voit, le champ d'intervention

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en adaptant notre ordre juridique national pour y intégrer les principes, les missions et les structures du Parquet européen, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui marque l'aboutissement d'une évolution, que l'on peut assurément considérer comme majeure, de la coopération judiciaire européenne. En effet, celle-ci va désormais sortir du champ exclusivement intergouvernemental qui était le sien jusqu'à maintenant. Pour la première fois, une instance européenne disposera de compétences judiciaires propres en matière pénale.

Fraudes massives à la TVA, corruption, détournement de fonds publics, abus de confiance, blanchiment d'argent ou encore délits douaniers pourront dès lors entrer dans le champ de compétence du Parquet européen, si toutefois ils affectent les recettes de l'Union européenne ou ses programmes de dépenses, tels que les fonds structurels ou les subventions agricoles. Il est vrai que, dans ces domaines, les performances des différents pays européens en matière d'enquêtes et de poursuites restent à ce jour pour le moins contrastées. Mais surtout, les outils déployés jusqu'à présent pour améliorer la coopération entre États membres n'ont pas, malgré leurs réels mérites, permis d'endiguer de manière satisfaisante le développement de certaines fraudes, et tout particulièrement celles faisant appel à des montages transfrontaliers complexes. Le cas de la fraude à la TVA intracommunautaire est sans aucun doute le plus parlant et le plus préoccupant. Le manque à gagner pour les finances de l'Union européenne, et à plus forte raison pour celles des États, est énorme. Ce sont ainsi à 60 milliards d'euros qui se volatiliseraient chaque année en Europe, principalement du fait de groupes criminels organisés, dont certains entretiennent par ailleurs des liens avec le terrorisme et contribuent à son financement.

pour renforcer, mais aussi homogénéiser, la réponse pénale apportée aux délits financiers affectant les intérêts de l'Union européenne. La création d'un Parquet européen répond clairement à cet objectif, notamment dans sa dimension transfrontalière. À cet égard, sa capacité à mener des enquêtes dans plusieurs États membres simultanément et le fait que les éléments de preuves qu'il y recueillera pourront être admis par toutes les juridictions nationales me paraissent représenter des avancées absolument essentielles. L'innovation que constitue le Parquet européen n'est pourtant pas allée sans susciter de longs et vifs débats, car, pour reprendre les termes de l'avis du Conseil d'État, si elle n'est pas contraire aux exigences de notre Constitution, son instauration touche aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. Les atteintes à ce principe, qui constitue le socle fondamental de l'application du droit pénal, me semblent cependant avoir été correctement circonscrites, notamment grâce à l'action du Sénat, qui a pleinement joué son rôle de gardien du principe de subsidiarité. Cela a été dit, le Sénat le Sénat a été à l'origine, avec treize autres assemblées parlementaires européennes, du déclenchement d'une procédure de « carton jaune » à l'encontre de la proposition initiale de la Commission européenne. développait une vision excessivement centralisée du Parquet européen, incarnée par la figure d'un procureur unique disposant d'une compétence exclusive pour diligenter des enquêtes dans toute l'Union européenne. Le compromis finalement trouvé, qui assure notamment sa structure collégiale et, au travers des procureurs européens délégués, son ancrage dans les structures et l'ordre juridiques des États membres, apparaît à la fois équilibré et réaliste. Ainsi, si la définition de la politique pénale et la supervision des affaires s'effectueront au niveau européen, les enquêtes seront conduites dans les États membres par des magistrats nationaux, les jugements seront prononcés par les juridictions nationales selon le droit national en vigueur et les éventuels conflits de compétence seront réglés par les autorités nationales. Cette intégration du Parquet européen dans la réalité juridique de chaque État membre était non seulement indispensable au regard du principe de subsidiarité, mais aussi impérative pour permettre au projet d'aller jusqu'à son terme. Elle n'en rendra pas moins nécessaire de rester vigilants quant à la bonne articulation opérationnelle du Parquet européen avec les juridictions françaises. L'étude d'impact qui accompagne le projet de loi indique qu'une centaine de dossiers tout au plus seraient susceptibles de relever chaque année de sa compétence. Si ce nombre relativement faible ne devrait pas entraîner de bouleversement fondamental dans l'organisation de la justice, le dispositif mis en place, notamment autour des prérogatives du procureur européen délégué, vient en revanche bousculer quelque peu l'ordonnancement traditionnel de notre cadre procédural. Il conviendra donc, dans les années à venir, d'observer attentivement la manière dont le Parquet européen exercera concrètement ses missions. C'est également la raison pour laquelle il me semble il me semble particulièrement prématuré d'appeler d'ores et déjà à l'extension de ses compétences, notamment à la lutte contre le terrorisme, matière éminemment sensible et délicate. Nous Nous n'y sommes pas favorables, bien que la Commission européenne et le Président de la République la souhaitent. J'observe d'ailleurs que, ces dernières années, l'Union européenne a

je crois qu'il nous faut rester prudents sur les missions supplémentaires qui pourraient éventuellement lui être confiées à l'avenir. Pour l'heure, il doit surtout faire la preuve de son efficacité et de sa plus-value dans la lutte

concentrons-nous avant tout sur la réussite de cette initiative majeure pour le développement d'une Europe capable de mieux protéger ses intérêts et de lutter plus efficacement contre la criminalité. La parole

La cheffe du Parquet européen pourra révoquer les PED pour des raisons disciplinaires. Enfin, les États membres ne pourront, à leur niveau, lancer de poursuites disciplinaires

territoires, où l'on s'inquiète de la désertification de certaines zones rurales, où certains citoyens ont l'impression d'une bulle parisienne déconnectée des

équitable figure le respect du principe du contradictoire, corollaire indissociable des droits de la défense. Ce principe vise à assurer l'information des parties sur les éléments de fait et de droit de l'affaire. Sont concernés ici l'assistance d'un avocat, la communication du dossier ou encore le mode de preuve utilisé. La chambre criminelle de la Cour de la cassation a par ailleurs affirmé le caractère absolu du respect du principe du contradictoire

a précisé les droits des personnes mises en examen, placées sous le statut de témoin assisté ou s'étant constituées parties civiles dans le cadre d'une instruction conduite par le procureur européen délégué.

Selon l'article 6 du règlement du Conseil du 12 octobre 2017, « le Parquet européen est indépendant ». L'ensemble de ses membres, parmi lesquels les procureurs européens délégués, ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune personne extérieure au Parquet européen, d'aucun État membre de l'Union européenne, ou d'aucune institution, d'aucun organe ou organisme de l'Union. l'Union. Les États membres de l'Union européenne [ ...] respectent l'indépendance du Parquet européen et ne cherchent pas à l'influencer dans l'exercice de ses missions. » Or l'article L. 228 du livre des procédures fiscales limite le pouvoir du procureur européen délégué, puisqu'il rend irrecevables « les plaintes portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux [cinq premiers] alinéas du I [ ...] déposées par l'administration à son initiative, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales

de ce débat : « Le verrou de Bercy bloque toute la chaîne pénale. Il empêche la variété des poursuites et constitue un obstacle théorique, juridique, constitutionnel et républicain, en plus d'être un handicap sur le plan pratique. » Le débat n'est donc pas définitivement clos,

55.

? « Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. « Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. » La constitution

premier est la condition de résidence habituelle sur le territoire français des auteurs de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité.

lorsqu'ils se trouvent en France. Ce serait la moindre des choses que d'en décider ainsi et de l'inscrire dans la loi, car ces criminels sont les pires qui soient.

En matière d'atteintes à l'environnement, il faut bien distinguer, comme le fait le rapport intitulé « Une justice pour l'environnement », les conflits environnementaux du quotidien des affaires à

L'histoire mondiale nous a malheureusement enseigné que des atteintes irréversibles à des écosystèmes ont eu des conséquences massives et très graves sur des populations entières, au point de mettre en question leur avenir sur leur territoire- je pense, par exemple, à l'emploi de l'agent orange au Vietnam. De telles atteintes peuvent affecter indirectement la santé de citoyens français, par migration de substances dangereuses par exemple. Il ne me semble dès lors pas disproportionné de réfléchir aux moyens de rendre nos juges compétents

Il s'agit toujours de permettre que les juridictions françaises soient compétentes pour juger les personnes résidant habituellement sur le territoire de la République qui auraient commis, à l'étranger, un crime ou un délit en bande organisée accompagné d'une atteinte à l'environnement. Le droit en vigueur prévoit que des poursuites sont possibles pour des faits commis à l'étranger, en cas de crime contre l'humanité ou de crimes de guerre, à condition qu'aucune juridiction nationale ou internationale ne demande l'extradition de la personne suspectée. Nous avons conscience

nécessiter des démarches diplomatiques conduites conjointement par le ministère de la justice et celui des affaires étrangères. Ce n'est donc que le début d'une réflexion à mener collectivement.

Notre commission des lois connaît les réserves de l'exécutif sur ce point et ces différents votes n'ont pas permis de convaincre l'Assemblée nationale.

les juridictions françaises, de se saisir d'une rupture de barrage en Chine ou d'une infraction en matière de biodiversité commise

ce sujet. Je rappelle que cette loi a modifié la compétence quasiment universelle de la France pour juger des génocides, crimes contre l'humanité et crimes et délits de guerre commis à l'étranger. Comme le Sénat l'avait proposé, elle a introduit la référence expresse aux génocides, crimes contre l'humanité et crimes et délits de guerre, en lieu et place d'un simple renvoi à la compétence de la CPI. Elle a également mis fin à la condition de double incrimination pour les crimes de génocide. Elle a aussi introduit la possibilité, en cas de classement sans suite, de former un recours devant le procureur général, lequel devra statuer après avoir entendu le requérant.

toute personne de passage en France pourrait faire l'objet de poursuites. Dès lors, même si le dispositif de l'amendement tend à maintenir le monopole des poursuites du parquet, il est à craindre que des associations n'adressent à ce magistrat des demandes médiatisées de poursuites en cas de visite en France de représentants d'États étrangers qu'elles accuseraient d'avoir commis tel ou tel crime contre l'humanité. Même si le procureur devait rejeter ces demandes, de telles pratiques pourraient être source de polémiques ou d'attentes difficiles à satisfaire et seraient susceptibles d'affecter l'action diplomatique de la France.

de la convention de l'ONU du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à l'unanimité. La jurisprudence de la Cour internationale de justice a établi que l'interdiction du génocide

rectifié, octroyer à la France une compétence quasiment universelle pour l'ensemble des infractions au code de l'environnement ne me paraît pas envisageable, pour plusieurs motifs. D'abord, décider de cette compétence quasiment universelle de manière unilatérale serait contraire au principe de la souveraineté des États. Il convient de rappeler qu'une telle compétence ne peut compétence ne peut résulter que de conventions internationales et qu'elle est, à ce jour, limitée aux crimes d'une extrême gravité, susceptibles d'être réprimés indépendamment des considérations de frontières ou de nationalité, parce qu'ils heurtent l'humanité dans son entier- je pense ici, évidemment, aux crimes de génocide, aux crimes de guerre, de tortures, etc.

question de la légitimité de la France à engager des procédures dépourvues de lien nécessaire avec notre pays, l'effectivité de celles-ci n'apparaît aucunement garantie dès lors que l'établissement de la preuve d'atteintes à l'environnement requiert notamment de procéder à des enquêtes sur les lieux où les faits ont été commis. En revanche, la lutte contre les atteintes à l'environnement à l'échelle mondiale nécessite

commises par les réseaux de délinquance et de criminalité organisée peuvent déjà faire l'objet d'une répression par les juridictions françaises, dès lors que l'un des faits constitutifs des infractions

par rapport aux autres dispositions du code de procédure pénale relatives à la compétence des tribunaux français en matière de répression des crimes internationaux. Je connais la position du Quai d'Orsay que vous relayez,

dans le cadre du mandat d'arrêt européen pour les infractions les plus graves, telles que le terrorisme, le trafic d'armes et la traite des êtres humains. Par conséquent, notre position me paraît fondée. J'espère que nous obtiendrons un jour satisfaction.

justice pour l'environnement » fait en effet état du manque de moyens d'enquête pour lutter contre les atteintes

doit évoluer afin que l'on puisse sanctionner les grandes entreprises qui tirent profit des infractions qu'elles commettent. Il faut tenir compte de ce caractère lucratif. Si les sanctions prévues par le code de l'environnement peuvent être multipliées par cinq en vertu de l'article 131-38 du code pénal, elles ne sauraient être suffisamment dissuasives pour les entreprises

lorsqu'ils constatent que l'atteinte à l'environnement permet d'espérer un gain supérieur au maximum de l'amende encourue, comme le recommande le rapport remis par le CGEDD justice en octobre dernier. Un tel dispositif s'inspire des sanctions prévues en matière de pratiques commerciales trompeuses. Le lien entre l'infraction et le chiffre d'affaires garantit la constitutionnalité de la mesure. Enfin, cet amendement tend à mieux tenir compte, de la directive du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement, qui dispose que les États membres doivent prévoir des peines effectives, proportionnées et dissuasives. Mes chers collègues, si la réparation des dommages causés à l'environnement est importante, la prévention l'est tout autant ! Quel est l'avis de la commission

souhaite modifier l'échelle des peines en matière de droit de l'environnement. Or traiter de l'échelle des peines est un exercice extrêmement complexe : il faut tenir compte de nombreuses dispositions administratives, de modalités d'amende, d'interdictions d'exploitation

Quelques chercheurs ont entendu l'appel du président Macron, mais Nicolas Hulot décide de quitter le navire, en raison d'un écart trop grand entre les discours et les actes. De la grande histoire à la petite, tout illustre le décalage entre les objectifs affichés et les petits pas accomplis grâce à la politique environnementale du Gouvernement. Les attentes sont pourtant fortes. Une partie de la jeunesse se mobilise et se radicalise, dans le courant, notamment, du mouvement Extinction Rebellion. Voilà quelques jours, plus de 1 000 scientifiques ont signé un appel à la mobilisation, en incluant la désobéissance civile. D'autres D'autres mouvements moins radicaux, mais tout aussi profonds, impriment encore l'opinion. Je pense ici à la plus belle réussite de l'exécutif en matière environnementale, à savoir la création de la Convention citoyenne pour le climat. Audacieuse sur la forme et dans ses objectifs, cette innovation institutionnelle soulève beaucoup d'espoirs. Madame la ministre, avez-vous pris en considération dans vos travaux, ces derniers mois, cette convention citoyenne qui travaille sur des sujets de justice climatique. Des députés sont allés parler d'écocide avec ces citoyens. Je ne sais pas si la convention se montrera plus ouverte à cette innovation juridique que la majorité sénatoriale ne l'a été ; j'espère que oui. On peut imaginer aussi que ces citoyens feront des propositions en termes de hiérarchie des peines en matière de délinquance et de criminalité environnementales, de moyens à la disposition de la justice. Quelle est votre opinion, madame la ministre, sur ces sujets ?

Faute de réponse satisfaisante, nous jugeons préférable de renvoyer à plus tard nos débats sur ces sujets, pour ne pas court-circuiter les travaux de cette utile Convention citoyenne

complexes, multiformes et trop peu sanctionnés. La biodiversité et le vivant n'ont jamais été autant menacés. L'arsenal législatif, pénal et répressif doit donc être porté à la hauteur des défis écologiques, pour la survie même de notre humanité.

d'une telle procédure et à la possibilité de mesures de réparation ou de compensation environnementale. Pour autant, nous restons dubitatifs, craignant que cette transaction n'ouvre la voie à une justice d'exception, sans procès ni droits de la défense ; une justice externalisée, idéale pour ne pas trop abîmer l'image des entreprises.

de doter ces structures de moyens spécifiques ; l'idée est simplement de nommer des référents pour les contentieux environnementaux au sein des juridictions existantes. Les juges ne s'y sont d'ailleurs pas trompés : ils demandent en priorité une

ont encore de beaux jours devant eux la création d'un nouveau mécanisme transactionnel pour régler les contentieux environnementaux les plus graves et la mise en place de juridictions spécialisées au sein des cours d'appel pour traiter de ces mêmes contentieux.

Deux mécanismes transactionnels permettent aujourd'hui de traiter les contentieux relevant du code de l'environnement. Grâce à la transaction et la composition pénales, près de 80 % des cas sont réglés en évitant la lourdeur d'un procès. Or transiger n'est aujourd'hui possible que pour les affaires les moins graves. Est-on sûr, dans ces conditions, que la nouvelle convention judiciaire créée à l'article 8 permettra de régler beaucoup de nouveaux cas ? Avons-nous une estimation du nombre d'affaires qui pourraient être réglées par le biais de la CJIP environnementale ?

Bien sûr, transiger permettra d'aller plus vite et de réduire des délais de jugement qui peuvent parfois atteindre près de trois ans aujourd'hui. Mais le vrai remède n'est pas de multiplier les mécanismes alternatifs

Ainsi, la loi portant création de l'Office français de la biodiversité a renforcé les pouvoirs et les prérogatives des inspecteurs de l'environnement.

Notre rapporteur, qui est assez dithyrambique à propos de cet outil qu'il juge « ultra-puissant », n'est pas suivi par le Syndicat de la magistrature, par exemple, qui considère que l'utilisation de la transaction résulte d'une conception économique de la justice, particulièrement étrangère à notre culture juridique, et que le coût financier de la commission d'une infraction pourrait être intégré par les sociétés comme n'importe quel coût, sans effet dissuasif. De plus, selon ce même syndicat, la CJIP ouvre la possibilité d'une négociation entre le procureur et l'entreprise poursuivie dans un contexte où le rapport de force risque d'être fortement déséquilibré au profit des entreprises, bien conseillées, et au détriment de l'autorité judiciaire, aux moyens plus limités. Le Syndicat de la magistrature évoque aussi une justice à deux vitesses et constate que cet outil pourrait ne pas être assez dissuasif.

on a perdu un peu d'argent, on en récupère ... Ce n'est pas très grave : « Plaie d'argent n'est pas mortelle. » Madame la ministre, vous avez parlé vous-même tout à l'heure de hisser notre organisation judiciaire à la hauteur des attentes de nos concitoyens.

obligation. La justice tord le bras de la personne morale, par exemple de l'entreprise qui commet des dégradations de l'environnement. Celle-ci se soumet à la procédure, fait preuve de bonne volonté ; on la surveille pendant un certain nombre d'années, en lui accordant un délai pour se mettre en situation

aux mêmes procédures judiciaires. Or les procédures ordinaires sont garantes non seulement des droits de la défense, mais également de l'ensemble des règles afférentes aux procès. L'expérience en matière fiscale devrait nous servir de leçon. En effet, c'est bien une convention judiciaire d'intérêt public qui a permis à la banque HSBC, mise en cause dans une affaire de blanchiment de fraude fiscale, de s'en sortir avec une simple amende de 300 millions d'euros.

Et vous voulez étendre ce dispositif aux délits environnementaux ! Nous n'y sommes bien sûr pas favorables. Nous demandons donc la suppression de cette mesure qui, sous couvert de rendre la justice avec célérité, remet en cause tous les principes d'une procédure équitable.

que l'arsenal répressif soit complété. Nous souhaitons enfin que les moyens humains de la police de l'environnement et de la justice soient renforcés. Sinon, aucune avancée en matière de justice environnementale ne pourra réellement être réalisée. La

est critiqué en matière financière, certains dénonçant un moyen d'acheter son innocence financière. De façon générale, ces conventions s'inspirent du système judiciaire et affaiblissent la place de l'autorité judiciaire dans le système pénal. Un tel dispositif n'est pas satisfaisant en matière environnementale, parce qu'un préjudice environnemental est plus difficile à évaluer qu'un préjudice financier. De même, la réparation du préjudice environnemental est parfois impossible, alors qu'elle est toujours possible en matière financière. Le parallèle établi ne nous semble donc pas totalement pertinent. En outre, ce dispositif pourrait fragiliser les PME au regard des grands groupes, dès lors que, faute de conseil juridique équivalent, elles se montreraient plus vertueuses que ces derniers, incités quant à eux à acheter un droit à polluer. Il faudra de toute façon procéder à une fine évaluation de ce dispositif s'il doit être mis en oeuvre.

C'est pourquoi nous considérons que, si le texte devait être maintenu en l'état, il conviendrait que ces conventions soient largement rendues publiques. Comme l'exigeait le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi, le dispositif proposé prévoit déjà que l'ordonnance de validation, le montant de l'amende d'intérêt public et la convention elle-même soient publiés sur les sites internet du ministère de la justice, du ministère chargé de l'environnement et de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise sur celui de l'établissement public de coopération intercommunale auquel ladite commune appartient. Tout cela va dans le bon sens, mais ne nous semble pas suffisant. Aussi proposons-nous tout simplement, au travers de cet amendement, que la publicité de ces nouvelles transactions environnementales soit renforcée

la convention et son contenu dans son rapport annuel. Cela permettrait d'aller au bout de la logique voulant que cette convention constitue,

est à M. Jérôme Durain. Avec cet amendement, nous souhaitons aller au bout de la logique proposée. Trop longtemps, nous nous sommes reposés sur l'idée selon laquelle les êtres humains étaient assez intelligents et raisonnables pour maîtriser eux-mêmes leurs dérives et préserver la planète. Une telle logique témoigne d'un orgueil démesuré ; elle nous a condamnés trop longtemps à l'inaction en matière environnementale. Le groupe socialiste et républicain entend rompre ce cercle vicieux. L'objectif est de poursuivre et de punir les délits, mais aussi les crimes les plus graves qui portent atteinte de manière irréversible à la « sécurité de la planète », pour reprendre les mots de Mireille Delmas-Marty. Il s'agit de poser les bases d'un droit pénal de l'environnement, permettant de lutter rigoureusement contre la criminalité environnementale et de punir sévèrement les auteurs de ces actes. Le Sénat a su, par le passé, être précurseur sur les questions environnementales, notamment en faisant adopter la notion de préjudice écologique, grâce à une proposition de loi déposée par Bruno Retailleau. Il s'agit maintenant d'aller plus loin dans le combat pour la préservation de la planète. C'est pourquoi notre groupe souhaite étendre le dispositif de l'article 8

« Une Justice pour l'environnement », il existe déjà, au sein des juridictions, des référents pour le contentieux de l'environnement, créés par la circulaire du 23 mai 2005. Cependant, comme le souligne ce même rapport, les recommandations de cette circulaire n'ont pas été suivies, faute de moyens

des autres agents et gardes que les inspecteurs de l'environnement ou les forces de police générale. Les gardes particuliers assermentés, notamment, sont des acteurs de proximité incontournables pour la dissuasion et sont habilités à la police des déchets.

comme des acteurs de la police de l'environnement, notamment en matière de chasse et de pêche. Cet article « chapeau » permettra également à l'Office français de la biodiversité de mettre en place des partenariats avec les gardes particuliers assermentés structurés en association.

les modifications proposées ne me paraissent pas opportunes, en particulier celles qui sont relatives à la possibilité, pour les gardes particuliers, d'adresser des amendes forfaitaires.

de présenter un amendement qui vise à introduire un droit d'évocation des affaires au bénéfice du parquet national financier, en matière de traitement des dossiers de fraude fiscale, sans remettre bien sûr en cause le principe de la compétence concurrente. Ce droit d'évocation, qui serait exercé de la procédure de concertation avec les parquets territorialement compétents, permettrait au PNF de mieux définir sa compétence, sur la base d'un principe de subsidiarité reposant sur des critères objectifs du fait de la technicité et de la complexité des investigations et des règles juridiques applicables. Il permettrait également de favoriser un traitement harmonisé des affaires similaires. Dans sa communication

et que la compétence de la juridiction territorialement la plus étendue l'emporte sur celle de la juridiction dont le ressort territorial est plus limité. Or le PNF est une juridiction spécialisée

à l'environnement. Lors de nos précédentes discussions, il a été dit que l'opportunité du dispositif de cet amendement n'était pas évidente. Certes, son périmètre pourrait être restreint aux atteintes les plus graves, mais cela nécessiterait un important travail d'inventaire de long terme. De nombreuses observations nous ont poussés à le redéposer. Il s'agit pour nous d'accélérer la prise de conscience sur la nécessité de renforcer les moyens d'enquête dévolus à la poursuite des infractions environnementales. Le rapport

compte tenu de la sensibilité accrue de nos concitoyens à ces questions. Comme il est souligné dans ce même rapport, « il n'y a pas de police efficace sans renseignement. Ce constat est particulièrement vrai pour rechercher et analyser les signaux faibles des atteintes à l'environnement. » Les moyens prévus à l'article 706-73 du code de procédure pénale pourraient permettre de repérer ces signaux faibles.

qui s'imposera un jour ou l'autre du fait de la multiplication des recours.

le crime de violence sexuelle sur enfant, en prévoyant que tout acte de pénétration sexuelle par une personne majeure commis sur une personne mineure de 15 ans est un crime de violence sexuelle sur enfant, puni d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle, la tentative étant punie de la même peine. Cet amendement tend à compléter la présomption de contrainte induite par l'écart d'âge prévue à l'article 222-22-1 du code pénal. Les travaux menés par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement son avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles, ont montré la nécessité de fixer un seuil d'âge en deçà duquel le non-consentement de la victime mineure

que nulle pénétration sexuelle ne saurait être involontaire. Le Conseil national de la protection de l'enfance recommande d'instaurer une infraction criminelle spécifique posant l'interdiction absolue, pour tout majeur, de commettre un acte de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans.

à la nouvelle donne environnementale. Il s'agit en particulier d'adapter la notion de mise en danger de la vie d'autrui, en prenant en compte une dimension future, et d'étendre cette

totalement notre approche pénale des atteintes à l'environnement et à changer de paradigme. Cet amendement tend donc à explorer une nouvelle piste d'adaptation

: La parole est à M. Jérôme Durain. Dans ce projet de loi, des solutions pour lutter contre les atteintes à l'environnement sont présentées, mais elles nous semblent- ce n'est pas une critique -bien insuffisantes et incomplètes. C'est pourquoi le groupe socialiste, à défaut d'avoir pu échanger davantage sur l'article 8 et de le rendre plus opérant, propose un dispositif global : organisation judiciaire, délits et infractions, nous vous proposons de mener de nouveau le débat sur la reconnaissance du crime d'écocide. Il s'agit de poser les jalons d'un droit pénal de l'environnement permettant de lutter frontalement contre les crimes qui menacent la planète, en introduisant, dans notre arsenal juridique, l'incrimination d'écocide. Cette nouvelle incrimination s'inscrirait dans le prolongement direct de la Charte de l'environnement, qui programme, dans son préambule, que « l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ». La Cour pénale internationale place les atteintes graves à l'environnement à la même hauteur que le terrorisme ou la traite des êtres humains et invite le législateur national à légiférer. Trop souvent, on nous rétorque : « Pas ici, pas maintenant », mais le contexte actuel de prise de conscience collective face aux atteintes à l'environnement nous oblige à développer notre arsenal législatif, pour créer un véritable droit pénal environnemental. Le Gouvernement a d'ailleurs admis à plusieurs reprises que, pour l'heure, il n'existait pas de dispositif permettant de sanctionner à leur juste mesure les atteintes les plus graves à l'environnement. Ce projet de loi est donc le bon véhicule législatif pour le faire. En matière de protection de l'environnement et du climat, il faut que nous soyons courageux, comme la France a pu l'être en d'autres périodes en matière de consécration des droits de l'homme. Nous avons la possibilité de devenir des pionniers de cette lutte contre la criminalité environnementale. Ouvrons la voie à des changements à l'échelon européen et international

En premier lieu, l'élément matériel du crime d'écocide ne paraît pas satisfaire à l'exigence constitutionnelle de clarté et de précision de la loi pénale, d'autant qu'il s'agirait ici, M. le rapporteur vient de le rappeler, d'une qualification criminelle. La définition du crime d'écocide est construite sur le modèle du crime de de génocide, puisqu'elle fait référence à l'exécution d'une action concertée tendue vers un but déterminé. Néanmoins, le crime d'écocide ne se définit que par les conséquences qu'il entraîne sur l'environnement ; il ne fait définit que par les conséquences qu'il entraîne sur l'environnement ; il ne fait aucune référence au comportement de la personne incriminée, comportement de nature à porter atteinte à l'environnement ou à la santé des personnes. En second lieu, s'il s'agit de réprimer au niveau international les atteintes graves à l'environnement, comme vous l'évoquez dans l'objet de votre amendement, l'adoption d'un corpus juridique de niveau international me semble être un

ainsi libellé : La parole est à M. Joël Labbé. L'éparpillement des infractions au sein de nombreux codes et la définition des infractions en fonction du non-respect d'une décision administrative entravent l'efficacité de la réponse pénale en matière environnementale.

du droit pénal de l'environnement, qui apparaît inféodé à la police administrative ». Il souligne par ailleurs la grande technicité de ce droit exigeant la démonstration d'un résultat dommageable souvent difficile à établir et propose la création d'une infraction générique d'atteinte volontaire à l'environnement, objet du présent amendement. La Conférence nationale des procureurs de la République se serait également prononcée en ce sens. La définition de l'infraction retenue dans l'amendement que nous proposons s'inspire en partie de l'article 326 du code pénal espagnol et de l'article L. 173-3 du code pénal français, qui sanctionne le non-respect d'une mise en demeure de l'administration ayant provoqué une dégradation substantielle de la faune, de la flore, de la qualité de l'air, du sol ou de l'eau. L'article 410-1 du code pénal reconnaît l'équilibre du milieu naturel et de l'environnement de la France au titre des intérêts fondamentaux de la Nation. Par une décision n° 2019-823 le Conseil constitutionnel a jugé que « la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains constitue un objectif de valeur constitutionnelle » et que sa préservation devait être recherchée « au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ». Ces considérations justifient de placer, comme l'évoque le rapport précité, ce nouveau chapitre au sein du titre I du livre IV du code pénal relatif aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.

auquel vous faites référence, la définition de la dégradation substantielle de la qualité de l'air est une définition administrative. Or l'amendement que vous proposez vise à créer un délit reposant sur cette dégradation substantielle de l'air. Cela suppose que le juge pénal,

Le caractère non intentionnel de nombreuses infractions environnementales et la difficulté de démontrer les atteintes à l'environnement expliquent en partie l'insuffisance de la réponse pénale, alors que les conséquences peuvent être graves pour l'environnement et la santé. Cet amendement vise à inciter les entreprises à la prévention des conduites à risque, grâce à la création d'un délit spécifique de mise en danger de l'environnement, attendu par les associations environnementales et préconisé par le rapport du CGEDD et de l'IGJ, sans pour autant avoir fait l'objet de propositions de rédaction. Ce délit sanctionnerait de deux ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende « le fait d'exposer directement ou indirectement la faune, la flore, la qualité de l'air, du sol, du sous-sol ou de l'eau, ou l'équilibre des écosystèmes à une dégradation substantielle par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, le règlement ou un acte administratif individuel ». L'ajout des actes administratifs individuels permettant de caractériser l'infraction est essentiel, puisque le droit pénal de l'environnement repose en partie sur le non-respect de décisions administratives. Il vise donc à sanctionner des comportements délibérés faisant peser un risque à l'environnement.

ne paraît pas correspondre à l'exigence constitutionnelle de précision de la loi pénale ; on en revient toujours à ce point. Le délit que vous proposez réprime le fait d'exposer l'équilibre des écosystèmes

ne se caractérise pas par son étendue, puisqu'il peut s'agir d'une mare à canards ou de quelque chose de beaucoup plus vaste. Il doit se caractériser par ses caractéristiques intrinsèques et s'applique donc à des échelles complètement différentes. Il me semble qu'il faudrait trouver sur ce point une écriture plus précise.

qui permettra d'éviter des erreurs d'interprétation ou de terrain. Actuellement, un garde qui est à la fois habilité aux titres de garde des fonds et des bois pour un même propriétaire, s'il verbalise dans le bois, peut relever l'identité du contrevenant, mais s'il s'agit de la même infraction de dépôts sauvages dans un milieu naturel non boisé, ne peut pas le faire. Ce frein ne fait que compliquer les actions de police menées par les gardes particuliers et les décourage de continuer à verbaliser. Cet amendement vise à harmoniser et à simplifier les actions de police judiciaire des gardes particuliers assermentés, la modification de l'article 29 du code de procédure pénale habilitant l'ensemble des gardes particuliers à cet effet. Jusqu'à présent, seuls les gardes particuliers des bois et forêts mentionnés à l'article L. 161-6 sont habilités à relever l'identité des personnes à l'encontre desquelles ils entendent dresser le procès-verbal. Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent ou le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale. En matière de lutte contre les atteintes à la biodiversité et de verbalisation des dépôts sauvages de déchets en milieu naturel, ce pouvoir de police permettrait aux gardes particuliers assermentés de toutes spécificités d'user, en lien avec l'officier de police judiciaire, à bon escient et objectivement, de ce droit de vérification d'identité des contrevenants ou délinquants. En l'absence d'harmonisation de cette prérogative, nombre de gardes particuliers dénoncent les infractions de dépôts sauvages de déchets par compte rendu adressé aux parquets. Ces derniers ne poursuivent que très peu les fautifs, sous prétexte qu'un compte qu'un compte rendu n'a pas de valeur probante, contrairement au procès-verbal de constatation d'infraction, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Mes chers

Cet amendement vise à faciliter les perquisitions, en permettant aux techniciens de l'environnement de participer aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction, sous la direction d'un officier de police judiciaire, sans avoir à prêter serment par écrit et à être inscrits sur l'une des listes des experts judiciaires. En effet, aujourd'hui, ces deux conditions sont requises et compliquent les enquêtes, alors que ces fonctionnaires et agents sont déjà commissionnés et assermentés à leur entrée en service.

différents dispositifs, pour lutter contre les atteintes à l'environnement et répondre à une réelle stratégie ambitieuse de protection de l'environnement.

dans le cadre d'une cosaisine, de participer aux perquisitions et aux saisies réalisées par les OPJ. Si je partage l'objectif de simplification évoqué au travers de ces deux amendements identiques, je suis favorable à ce qu'une autre solution rédactionnelle puisse être trouvée. Là encore, je pense qu'un tel travail pourra être réalisé au cours de la navette parlementaire.

Cet amendement vise à permettre, pour lutter contre le trafic international d'espèces sauvages et de déchets, l'échange d'informations et de documents et la coopération des inspecteurs de l'environnement avec les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne. En effet, ce n'est pas prévu par le droit actuel, alors que cette coopération permettrait une meilleure efficacité

des mesures relatives aux rejets volontaires d'hydrocarbures en mer par les navires, nous proposons de permettre l'immobilisation d'un navire ayant jeté ses eaux de ballast chargées d'organismes nuisibles et pathogènes dans les eaux françaises, dans l'attente du paiement d'un cautionnement. Avec un tel système, les responsables de l'infraction ne récupèrent leur caution qu'une fois déduits l'amende, les dommages, les intérêts et les frais de justice, ce qui garantit le paiement des amendes et la réparation des dommages. Ce dispositif permet une meilleure efficacité dans le recouvrement des amendes, comme cela se vérifie en pratique dans le cas des rejets volontaires d'hydrocarbures. En l'absence de cautionnement, les condamnations prononcées contre des capitaines et des armateurs de tels navires étrangers restent inexécutées. De récentes poursuites datant du mois de janvier 2020 devant le tribunal correctionnel de Rouen contre des capitaines et armateurs étrangers de différentes nationalités pour ces chefs d'accusation ont révélé cette lacune du droit. Notre amendement vise donc à y remédier.

la peine complémentaire de confiscation de la chose ayant servi ou été destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit me semble la piste la plus prometteuse. Le Gouvernement s'engage donc à examiner attentivement les situations dans lesquelles cette peine complémentaire de confiscation pourrait être plus facilement mobilisée pour dissuader les atteintes à l'environnement.

Cette proposition découle d'une préoccupation des avocats pénalistes. L'article 9 vise à déterminer les conditions dans lesquelles les officiers et agents de police judiciaire peuvent, en vertu d'une autorisation générale du parquet, faire procéder à des examens médicaux et psychologiques, avoir accès aux différents systèmes de vidéoprotection dans le cadre d'une enquête préliminaire. Il permet également aux de faire procéder, toujours sans autorisation du parquet, à des comparaisons d'empreintes ou de traces génétiques ou digitales. Il s'agit de s'assurer qu'il n'y a pas d'autorisation générale et systématique du parquet. Chaque procédure devrait continuer de faire l'objet d'une autorisation spécifique du procureur. Autoriser les OPJ à collecter et traiter des empreintes et traces génétiques ou digitales et à avoir accès aux différents systèmes de vidéoprotection sans autorisation préalable du procureur porte une atteinte disproportionnée à l'intégrité et aux droits fondamentaux de la personne physique mise en cause. L'obligation pour l'OPJ de se référer au procureur de la République est une garantie qu'il convient de maintenir dans le droit national. Jusqu'où irons-nous pour décharger les parquets afin de gagner du temps, faute d'un renforcement substantiel des moyens humains de nos juridictions ? Décharger le procureur de certaines tâches et missions ne doit pas conduire à la dégradation de la protection des droits fondamentaux, ces mêmes droits fondamentaux et constitutionnels

En outre, elles ne concernent que certains actes extrêmement fréquents dans les enquêtes ; M. le rapporteur les a évoquées. Enfin, les autorisations ne sont accordées que pour une durée de six mois. Il me semble que le texte initial présente un juste équilibre entre des considérations pratiques et la nécessaire surveillance par le parquet des actes accomplis par la police judiciaire.

outre une importante réforme de l'organisation judiciaire, la spécialisation de tribunaux désignés par décret pour juger dans l'ensemble du département de certaines matières civiles et de certains délits ou contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État. Pour la mise en oeuvre de la spécialisation, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort, après avis des chefs des juridictions concernées. Cette évolution intéressante a été insérée dans un nouvel article L. 211-9-3 du code de l'organisation judiciaire. Néanmoins, la spécialisation départementale ne couvre pas l'intégralité des problèmes qui se posent, notamment le cas de tribunaux dont les ressorts ne couvrent pas l'ensemble du département.

vise à corriger la rédaction de l'article L. 211-9-3 du code de l'organisation judiciaire, pour que la spécialisation couvre l'ensemble des ressorts de ces juridictions, et non plus l'ensemble du département.

à Mme Éliane Assassi. Au travers de cet amendement de repli, nous demandons que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur l'utilisation réelle de la procédure de convention judiciaire d'intérêt public dans le domaine de l'environnement. Par pragmatisme, nous souhaitons que les élus de la République disposent de données précises et fiables sur le nombre de conventions conclues chaque année, mais également sur le niveau des amendes et des réparations imposées. Quel est l'avis de

27. L'article 11, dont nous demandons la suppression, prévoit la création d'une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports lorsque les faits sont commis en état de récidive de certains délits ; j'y ai

ni disproportionné ni inefficace. En effet, la peine est mesurée dans son quantum et ne s'adresse qu'à un certain nombre de personnes. Par exemple, elle ne sera pas applicable aux mineurs de moins de 16 ans. Par ailleurs, la juridiction devra délimiter précisément les portions de réseaux de transport, en tenant compte, comme l'a dit M. le rapporteur, des contraintes de la vie familiale et professionnelle,

Ces zones sont celles où les ministres de la justice et de l'économie estiment, après avis de l'Autorité de la concurrence, que la création de nouveaux offices n'est pas utile. La procédure d'installation de nouveaux professionnels libéraux après appel à manifestation d'intérêt ne s'y applique donc pas. Au contraire, dans les zones d'installation contrôlée, le ministre de la justice peut rejeter une demande de création d'un nouvel office, après avis de l'Autorité de la concurrence. donc plus simple que, dans les zones où aucun besoin n'a été identifié au moment de l'élaboration bisannuelle de la carte des zones d'installation, la création d'offices soit désormais prohibée en principe, sauf décision contraire du garde des sceaux, prise après avis de l'Autorité, et à condition de ne pas porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu. Quel

que ce soit dans la version initiale du Gouvernement ou dans le texte issu des travaux de la commission, vise à garantir l'accès au droit et à la justice, en assurant une couverture du territoire par les notaires et les commissaires de justice.

disparaîtront, asphyxiés par cette hausse des cotisations retraite. « Afin d'éviter les hausses de cotisation pour les avocats les plus vulnérables » et « de préserver l'équilibre économique des cabinets d'avocats », le Gouvernement, sous votre plume, madame la garde des sceaux, explique avoir déposé un amendement visant à instaurer « un dispositif de solidarité géré par la Caisse nationale des barreaux français, Selon le Gouvernement, la hausse de cotisation serait prise en charge « pour les avocats dont le revenu serait inférieur à 80 000 euros ». Il faut se reporter au texte de l'amendement présenté par le Gouvernement pour comprendre que cette prise en charge serait faite par la CNBF elle-même

Le Gouvernement accepte ainsi que cette mission indispensable au bon fonctionnement de la justice soit tributaire du professionnalisme et de l'engagement des avocats envers les justiciables. Cela n'est pas possible ! Aussi, madame la garde -de vouloir s'attaquer à leur régime actuel de retraite, qui est autonome, équilibré, pérenne, solidaire et prévoyant. Le présent amendement vise donc à reconnaître cette profession, y compris dans ses droits en matière de retraite.

: lorsque la commission des lois émet un avis défavorable pour une raison technique, cela ne préjuge pas de la position qui sera prise par les uns et les autres,

il semblerait que le moment ne soit pas venu en cette fin d'après-midi.

Ensuite, sur la question des retraites, nous avions dès le départ des postulats qui étaient opposés. Nous souhaitions, car il ne peut pas en être autrement, que les avocats entrent dans le système universel des retraites. Ils ne le souhaitaient pas, pour des raisons que je puis raisons que je puis entendre, mais qui ne sont pas compatibles avec le projet ambitieux que nous portons. Il n'est pas possible qu'il y ait un système universel de retraite pour 66 millions de Français et un autre pour 70 000 avocats. Dans le le cadre de ce système universel de retraite, nous avons dit sans cesse que nous étions prêts à prendre en considération les spécificités

qui illustre les difficultés d'un système universel de retraite, compte tenu des spécificités d'un certain nombre de professions. À cet égard, les avocats sont un bon

que vous envisagez de discuter avec eux le respect du secret professionnel. En effet, nous sortons d'une audition de la commission des finances et du groupe de suivi sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, et la transposition de la directive européenne, qui doit entrer en application le 1 juillet prochain, pose des problèmes absolument terrifiants de respect du secret professionnel. En réalité, on va faire de l'avocat non seulement le complice, mais aussi le premier informateur des services fiscaux, au détriment de son client, quand bien même il ne serait pas au fait de la totalité de la situation fiscale de ce dernier. La directive n'étant pas encore transposée, elle relève pour le moment du domaine réglementaire.